Rémi Cardon, sénateur de la Somme

En application de l’article 28 de la Constitution, la session ordinaire de 2023-2024 est ouverte. Sénat a reçu communication de la liste des sénateurs proclamés élus le 24 septembre 2023. Acte est donné de cette communication.

pour la seconde fois, j’ai l’honneur de présider cette séance en vertu du privilège de l’âge. À ce titre, je voudrais vous livrer une recette

Plus sérieusement, mes premiers mots sont pour présenter mes sincères et chaleureuses félicitations à l’ensemble des sénatrices et des sénateurs nouvellement élus ou réélus dimanche dernier ; je leur souhaite la bienvenue au sein de notre assemblée. J’ai aussi une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui ne siégeront plus parmi nous, soit parce qu’ils n’ont pas souhaité se représenter, soit parce qu’ils n’ont pas été reconduits. Qu’ils soient remerciés de leurs actions constructives dans tous les domaines, de la qualité de leur travail et de leur participation à nos débats.

disait : « À l’Assemblée nationale, on tue avec le poignard. Au Sénat, on empoisonne avec le sourire. » Loin des turbulences du Palais-Bourbon, souvent soumis aux soubresauts de l’actualité, la Haute Assemblée reste un espace de stabilité dans nos institutions, où l’on sait que la politique, c’est l’art du compromis. le Sénat ne vit pas moins intensément le débat ; il a toujours su faire place à la confrontation et au respect des idées. Il est le garant de notre démocratie et fabrique la loi de façon plus subtile et peut-être plus réaliste. Nous sommes avant tout des parlementaires et, dans un régime qui l’est de moins en moins, le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques sont plus que jamais essentiels. part, je reste un partisan acharné du dialogue constructif, de la coconstruction des lois avec le Gouvernement et l’Assemblée nationale, où certains députés, malheureusement, ne comprennent pas toujours que ce qui leur reste de pouvoir réside dans le dialogue avec nous. C’est une manière de rendre le bicamérisme vivant, car celui-ci est un antidote à toute forme de populisme et d’extrémisme, ces maux qui menacent la cohésion sociale et la construction européenne. Les ingénieurs du chaos sont à l’œuvre ; il est urgent d’enrayer la machine à détruire la démocratie. Face à cette menace, il nous faut mobiliser en priorité les élus locaux, ceux qui sont en première ligne et que j’appellerais « l’armée de la République du quotidien se sentent parfois incompris ou délaissés, et nous sommes ici leurs représentants. Le rôle du Sénat est donc plus que jamais, en tant qu’assemblée des territoires, de relever les défis qui nous entourent la fracture territoriale, la perte d’autonomie fiscale, l’empilement des normes, la transition énergétique et la sécurité, entre autres. Je ne doute pas que la somme des talents, des compétences et des expériences que compte notre assemblée renouvelée apportera beaucoup à la fabrication de la loi et à la résolution de ces enjeux majeurs, avec ce « courage de la nuance » qu’évoquait Albert Camus, bien loin des facilités de l’outrance. Mes chers collègues, l’heure n’est plus à la mise en cause de l’existence du Sénat – Dieu merci ! –, bien au contraire. Tout le monde aujourd’hui en a pris conscience, lorsque l’une des deux assemblées boite ou vacille, l’autre apporte l’équilibre indispensable au bon fonctionnement de nos institutions. Par gros temps,

président. L’ordre du jour appelle le scrutin pour l’élection du président du Sénat. J’ai été saisi des candidatures

Conformément à l’article 2 du règlement, cette élection a lieu au scrutin secret à la tribune. Pour être élu au premier tour, un candidat à la présidence du Sénat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour, la majorité relative suffit. Je vous rappelle que les délégations de vote sont admises, mais que le délai limite pour la transmission des délégations de vote est désormais expiré depuis treize heures. La liste des délégations de vote a été régulièrement adressée à la présidence. Les sénateurs qui ont reçu une délégation pourront venir voter à l’appel soit de leur nom, soit de celui du délégant. J’invite nos deux plus jeunes secrétaires d’âge, Mme Mathilde Ollivier et M. Rémi Cardon, à superviser les opérations de vote. vote. Mes chers collègues, des bulletins de vote et une enveloppe ont été disposés sur votre pupitre. Vous serez invités à voter à la tribune en remettant votre enveloppe à la plus jeune secrétaire d’âge, qui la placera dans l’urne. Je vous rappelle que vous pourrez voter à l’appel de votre nom ou de celui de votre délégant.

être procédé à l’appel nominal de nos collègues, en appelant tout d’abord ceux dont le nom commence par une lettre tirée au sort il sera ensuite procédé à un nouvel appel des sénateurs qui n’auront pas répondu au premier appel de leur nom. Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera

voix. M. Gérard Larcher ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, je le proclame président du Sénat.

Je souhaite également remercier les secrétaires du bureau d’âge, fonction éphémère que j’ai exercée – c’était il y a quelques années C’est un moment un peu particulier. Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux collègues. Ils deviennent les héritiers et les porteurs du bicamérisme.

une période particulièrement noire, « l’État français », où le Parlement et la République avaient disparu. Mes chers collègues, le bicamérisme est indispensable à notre démocratie parlementaire. J’ai une pensée de gratitude pour celles et ceux qui ne siègent plus parmi nous aujourd’hui. Ils ont apporté au Sénat et au pays. Monsieur le doyen, vous avez eu, vous aussi, une pensée particulière pour eux. Permettez-moi de remercier très sincèrement celles et ceux qui m’ont témoigné leur confiance. Je m’engage à présider notre assemblée avec la légitimité que me donne la majorité, mais aussi dans le respect de vos diverses sensibilités. Je vous propose de n’avoir pour boussole que l’intérêt de notre pays et de poursuivre la construction du Sénat de demain. Je salue sincèrement Patrick Kanner, Cécile Cukierman et Guillaume Gontard, les présidents de groupe qui ont été candidats. Ils ont témoigné de la pluralité de notre assemblée. Je veux leur dire que je serai, comme hier, très attentif au respect des groupes minoritaires et d’opposition, comme d’ailleurs à chaque groupe politique et à chaque sénateur, où qu’il siège. Oui, il existe une manière particulière au Sénat d’exercer la fonction parlementaire. Être sénatrice, être sénateur, c’est faire vivre la démocratie, être au service de la République et des citoyens.

Nous incarnons plus que jamais ce pôle de stabilité, ce point d’équilibre que vous m’avez souvent entendu évoquer. Oui, je pense que le Sénat est plus que jamais au cœur de notre vie démocratique. Être sénatrice, être sénateur, c’est être autonome, libre et indépendant. C’est aussi se respecter les uns les autres. C’est donner à nos compatriotes le visage d’une assemblée où l’on débat, où l’on propose, où parfois l’on s’oppose, mais jamais dans le mépris, l’invective ou la violence. Mes chers collègues, il y a, me semble-t-il, une façon sénatoriale de faire de la politique : avec sérieux, calme et détermination. C’est la bonne méthode pour recoudre un pays fracturé, sans craindre de dire la vérité, même si elle dérange, et en ne reculant jamais devant l’obstacle. Forts de ces principes, nous devons imaginer et construire ensemble le Sénat de demain, pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens et des territoires, pour retrouver la confiance. Notre pays, qui souffre, qui doute, qui au fond n’a plus confiance, a besoin d’une assemblée attentive et – j’ose le dire – d’une assemblée presque affective à l’égard de nos compatriotes. Ces dernières années, j’ai sillonné le pays. J’ai rencontré de nombreux élus locaux et nombre d’acteurs économiques et sociaux. Vous le sentez bien, nous traversons une crise profonde aggravation des fractures territoriales, montée de l’abstention et des votes contestataires, dégradation de nos services publics et de la présence médicale, envolée de la dette publique et des déficits, montée des violences et des émeutes urbaines, inquiétude quotidienne face à l’inflation. La jeunesse est inquiète elle aussi, notamment face au défi climatique.

Le Président de la République a par deux fois, en 2017 et en 2022, annoncé son intention de procéder à une réforme des institutions. J’ai souhaité chaque fois que le Sénat soit dans l’anticipation. Notre groupe de travail transpartisan, qui se réunit depuis novembre 2022, formulera des propositions d’ici à la fin de cette année. Nous sommes prêts à envisager toute réforme à même d’améliorer le fonctionnement de notre démocratie, si elle permet de recoudre le pays, si elle permet au peuple de retrouver confiance en ses parlementaires, en ses gouvernants et en sa justice. et je le répète, notre Constitution ne se modifie pas en fonction des pulsions du moment.

Nous avons lutté contre le recours excessif aux ordonnances, qui dépossèdent le Parlement du débat et du droit d’amendement. La loi, pour retrouver sa force et son efficacité, doit obéir à quelques principes simplicité, lisibilité, efficacité ou encore subsidiarité. Il nous faut donc moins légiférer

L’annonce d’un projet de loi est trop souvent devenue un outil de communication… C’est vrai ! … pour les réseaux sociaux et les médias. Méfions-nous des lois de pulsion, à l’origine d’une inflation législative qu’il nous faut combattre.

« la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » – c’est l’article XV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. C’est ce que nous avons fait au cours de ces trois années, et c’est ce que nous ferons. Enfin, nous portons la voix des territoires. Nous sommes convaincus que la gouvernance verticale, la suradministration et l’hyperconcentration du pouvoir sont en partie à l’origine des maux dont souffre notre pays. Nous devons replacer les maires au cœur de la décision, gérer en proximité et imposer un nouveau souffle de décentralisation. Mais à une décentralisation forte, il faut un État territorial fort.

Le 6 juillet dernier, quinze propositions pour rendre aux élus leur « pouvoir d’agir » ont été publiées et adressées au Président de la République et à la Première ministre. simplification, l’autonomie fiscale et financière, le statut de l’élu, la relation entre les services de l’État et les maires, le logement et bien d’autres sujets encore.

En ces temps où l’équilibre institutionnel a été profondément modifié du fait de l’absence de majorité à l’Assemblée nationale, en ces temps où le fait majoritaire n’est plus, le Sénat a un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos institutions. Il est devenu le point d’équilibre d’une démocratie à la peine. Il est une assemblée qui assume ses différences et qui résiste à la désinformation, parfois alarmante, ainsi qu’à la « justice » expéditive des réseaux sociaux.

notre régime électoral [peut] nous empêche[r] de connaître les majorités cohérentes qui assurent, sans règles détaillées, la bonne marche du régime parlementaire

la démocratie représentative est fragile. Il faut en prendre soin. Veillons à l’image que nous projetons dans l’opinion. Faisons-la vivre en étant ouverts, disponibles et à l’écoute. Soyons attentifs au pouls de la société. À l’extérieur du pays naît un doute sur le rôle et le rang de la France dans le monde. Au cours de mes déplacements à l’étranger, j’ai rencontré nos compatriotes établis hors de France

Soyons attentifs aux puissances nouvelles qui émergent sur le continent africain et dans l’Indo-Pacifique, lesquelles bouleversent des équilibres qui semblaient durablement ancrés.

Ensemble, nous allons vivre trois années d’engagement au service des Français et de la République. Je crois profondément que le Sénat aura une responsabilité particulière pour mobiliser les forces vives de notre pays et pour faire vivre la démocratie. Nous devrons rester l’assemblée du débat apaisé, une assemblée responsable face aux défis qui se présentent, mais intransigeante chaque fois que les intérêts de la France l’exigent.

élément fort de notre culture ! J’attire votre attention sur l’importance de votre présence et de votre ponctualité pour la réalisation de la photographie officielle du Sénat dans l’hémicycle le jeudi 5 octobre,